je le reconnais volontiers : de prime abord, cette proposition de loi paraît séduisante. L’ouvrage, de Victor Castanet, a mis en exergue des défaillances importantes dans la gestion et le et le contrôle des Ehpad privés à but lucratif, qui recherchent de façon effrénée le profit au détriment de la qualité de vie des résidents. De même, la mission flash sur la gestion financière des Ehpad a montré que les établissements privés à but lucratif pratiquaient un prix moyen du séjour supérieur de 40 % au secteur public. De plus, le secteur des Ehpad rencontre des difficultés économiques d’une ampleur inédite. Elles sont dues aux tensions de recrutement, entraînant un plus faible niveau d’activité, d’activité, à la perte de confiance du public, à la suite de la crise du covid 19 et du scandale Orpea, ainsi qu’à un « effet ciseaux », entre la forte inflation des coûts et la moindre évolution des tarifs. Entre 2020 et 2023, la part des Ehpad déficitaires, tous statuts confondus, est ainsi passée de 27 % à 66 %. Dans ce contexte, on pourrait penser qu’une taxation des Ehpad privés lucratifs serait utile pour financer des mesures de soutien au secteur, d’autant plus que les besoins iront croissant au vu du vieillissement de notre population.

troisième du secteur, passé sous le contrôle d’un groupement d’actionnaires mené par la Caisse des dépôts et consignations. Alors que le secteur cherche à identifier des moyens pour stabiliser son modèle économique, cette proposition de loi semble peu opportune. D’autant plus qu’elle tend à ignorer certaines disparités territoriales, notamment en outre mer. En Guadeloupe, par exemple, l’offre d’hébergement en Ehpad est pourvue à 50 % par des structures privées à but lucratif. En attendant un rattrapage de l’offre publique en outre mer, ce que recommande le rapport d’information y taxer les Ehpad privés à but lucratif se révélerait contre productif, d’autant que les places manquent pour faire face au vieillissement accéléré de la population. Afin d’assurer la pérennité du secteur, il nous paraît plus efficace de soutenir et de mettre en œuvre les recommandations du rapport d’information. Parmi les propositions formulées par Solanges Nadille, Anne Souyris et Chantal Deseyne figurent la création d’une deuxième journée de solidarité pour financer la branche autonomie, l’instauration d’un plancher de revalorisation du tarif hébergement

votera contre cette proposition de loi. Cela ne signifie pas pour autant que nous signons un chèque en blanc aux Ehpad privés à but lucratif. Nous considérons qu’il est nécessaire de continuer à mettre en œuvre les mesures d’encadrement décidées par les gouvernements successifs de la majorité présidentielle, tout en évaluant leur efficacité. Tout d’abord, il sera

Il faudra ensuite s’assurer du respect des obligations de transparence renforcées dans les contrats de séjour des Ehpad. Enfin, nous devrons évaluer les mesures de prévention et de lutte contre les maltraitances, dont le respect de l’effectivité du droit de visite mettre en place une taxation sur un secteur en crise, qui limiterait encore les capacités d’hébergement, en particulier en outre mer, nous préférons poursuivre le travail d’encadrement pour rétablir la qualité et regagner la confiance des citoyens.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je tiens avant tout à saluer l’initiative de notre collègue Jean Luc Fichet. Ce texte nous permet de débattre d’un sujet qui nous concerne tous, car il symbolise le traitement que nous réservons à nos aînés et le soutien que nous offrons à ceux qui les accompagnent au quotidien. Cette question est d’autant plus prégnante que nous faisons face à un défi démographique majeur. D’ici à 2050, la France comptera près de cinq millions de personnes âgées de plus de 85 ans. Le vieillissement de la population va inévitablement augmenter la demande de solutions d’hébergement adapté. Il est donc crucial de préparer l’avenir dès maintenant, en renforçant nos Ehpad, en adaptant leur modèle économique et en assurant leur viabilité. Le récent rapport d’information de nos collègues Chantal Deseyne, Solanges Nadille et Anne Souyris rappelle combien la situation financière de ces établissements s’est fortement dégradée au cours des dernières années. Les Ehpad traversent aujourd’hui une période de crise les structures manquent de financement ; les conditions de travail y sont éprouvantes pour le personnel soignant ; leur coût est exorbitant pour les familles. Tous ces défis mettent à mal la dignité de nos aînés et de ceux qui les soignent. Nous ne pouvons pas ignorer cette réalité : trop souvent, les établissements souffrent de sous effectifs et les soins apportés ne sont pas à la hauteur de ce que méritent nos anciens. C’est une situation à laquelle nous devons faire face collectivement, avec responsabilité. Cette crise a des conséquences profondes sur la vie des résidents des Ehpad. Les scandales récents, tels que celui d’Orpea, ont mis en lumière des pratiques inacceptables qui vont à l’encontre du respect et de la dignité des personnes âgées. Ces dérives, bien que minoritaires, doivent être combattues. Elles ont rappelé l’importance de renforcer les contrôles, d’assurer une transparence totale et de faire de la qualité des soins une priorité. N’oublions pas non plus l’impact humain sur les soignants. Ces femmes et ces hommes engagés et dévoués travaillent dans des conditions difficiles, souvent épuisantes. Alors qu’ils sont le cœur battant de nos Ehpad, ils sont souvent sous payés et souffrent d’un manque de reconnaissance. N’est il pas essentiel de leur offrir des conditions de travail dignes, à la hauteur de leur engagement ? Pour cela, des investissements massifs sont nécessaires. Nous devons réformer le secteur de l’aide à la dépendance, améliorer le ratio personnel résidents et veiller à ce que les coûts pour les familles soient raisonnables. effet, la prise en charge de la dépendance ne saurait être un fardeau financier insupportable. Dans ce contexte, vouloir réformer le financement des Ehpad est une démarche tout à fait louable, et nous y souscrivons évidemment Pour autant, nous sommes plus réservés quant au « remède » proposé. Le texte de nos collègues vise en effet à créer une contribution additionnelle à la charge des Ehpad privés à but lucratif. Si j’en crois l’estimation faite par les services du ministère chargé des finances,

d’autant que le vieillissement de la population implique des besoins d’investissement dans les Ehpad qui pèsent notamment sur le secteur commercial. Il conviendrait aussi que nous abordions un jour le sujet des résidences autonomie et des résidences seniors privées, qui pourraient être fortement concernées par le problème de la rentabilité financière.

Je tiens à saluer l’initiative de notre collègue Jean Luc Fichet, que je remercie pour sa contribution sur un sujet qui nous touche tous de près ou de loin, celui du grand âge, de son accompagnement et de son financement. La gestion privée des Ehpad en France est devenue à juste titre un sujet de débat de premier plan. Alors que le secteur privé était quasiment absent de ce

Ces révélations ont mis en lumière la financiarisation du milieu consécutive à l’arrivée du secteur privé à but lucratif, suscitant inquiétudes et indignation quant à la qualité des soins et des services fournis aux personnes âgées. La sécurité et le bien être des personnes âgées sont au cœur des préoccupations de toutes les familles. Les faits révélés et dénoncés dans le cadre des

La médiatisation de ce sujet a ébranlé le système tout entier, et ce fut heureux. Elle a aussi plongé certains établissements dans une situation financière et budgétaire très dégradée.

Le maintien à domicile, qui appellerait du reste des politiques spécifiques plus abouties, doit être autant que possible recherché, mais, nous le savons, le nombre de nos aînés accueillis en Ehpad est appelé à aller croissant. Nous partageons le constat selon lequel les pouvoirs publics, sans doute pris de court par la financiarisation du secteur, n’ont pas réussi à le contrôler. Toutefois, le secteur privé reste nécessaire. Il doit apporter des garanties quant à la qualité de l’accueil de nos aînés

serait de réduire un peu plus les marges de manœuvre d’un secteur qui, en tout état de cause, est par trop affaibli. Depuis 2020, une situation conjoncturelle dégrade la rentabilité économique et la situation financière de ces établissements.

Alors que le secteur cherche plutôt à identifier des moyens de stabiliser son modèle économique, cette proposition de loi ne paraît pas apporter la garantie attendue. Même si l’on peut comprendre l’intention de ses auteurs, on peut douter de l’efficacité du dispositif

De moindres investissements ne feraient qu’accroître la pression pesant sur les secteurs privés à but non lucratif et public. Pour toutes les raisons que je viens d’invoquer, et malgré l’utilité de la démarche lancée par notre collègue Fichet, le groupe Union Centriste ne votera pas ce texte, considérant que le dispositif a plus de chances d’affaiblir le secteur que de lui apporter une solution pérenne. La parole

Poly. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je remercie mes collègues du groupe socialiste d’avoir inscrit ce texte à l’ordre du jour

Alors que 85 % des Ehpad publics sont actuellement en déficit, l’urgence est à une loi de programmation pluriannuelle sur le grand âge ; or un tel texte n’a toujours pas vu le jour. L’État doit prendre ses responsabilités, y compris à l’égard des départements, lesquels ne peuvent plus supporter des dépenses qui s’envolent. Les gouvernements successifs ont tous pris des engagements, sans jamais les tenir.

Face aux dérives du secteur privé lucratif, au manque d’attractivité des métiers, à la perte de confiance du public consécutive à la crise de la covid 19 et à la scandaleuse affaire Orpea, il y a urgence à revoir les modèles d’organisation et de financement des Ehpad.

nos yeux, cette taxation est la moindre des choses au regard des dérives liées à la financiarisation de la santé et des bénéfices réalisés sur le dos de nos aînés. définitive, la question n’est pas celle du niveau de profits réalisé par les établissements ; elle est celle de l’existence d’un secteur privé lucratif dans la santé et le secteur médico social.

proposition de loi constitue un petit pas sur le long chemin de la création d’un véritable service public de la perte d’autonomie. Pour l’ensemble des raisons que j’ai exposées, les sénatrices et sénateurs du groupe CRCE

Souyris. le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je tiens pour commencer à remercier le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain de nous permettre de débattre de la proposition de loi de notre collègue Jean Luc Fichet, que je salue. Les Ehpad font face à une crise sans précédent : déficit chronique insoutenable, métiers en extrême tension, investissement en berne, risques de fermeture pour cessation de paiements.

cette dernière année. Surtout, l’activité profitable des grands groupes privés lucratifs se fait au détriment de la sécurité sociale, des départements et de la justice fiscale. En effet, le budget des Ehpad se compose de trois parties, dont deux sont respectivement financées par les départements et par la sécurité sociale. Par ailleurs, les groupes privés optimisent leur profit la spéculation immobilière au détriment des usagers et des contribuables, comme l’a démontré notre collègue Raymonde Poncet Monge dans sa contribution au rapport sénatorial sur le contrôle des Ehpad. Entendu que les Ehpad privés commerciaux fonctionnent donc grâce à de l’argent public, il est normal qu’ils participent à notre effort collectif

des travaux de la mission que nous avons conduite ces derniers mois, nous avons compris que les Ehpad privés commerciaux prenaient en charge les hébergements les moins médicalisés, donc les plus rentables. J’ai donc proposé, dans notre rapport d’information, la création d’un cahier des charges pour les Ehpad commerciaux, afin que ceux ci prennent une juste part des places habilitées à l’aide sociale et des hébergements qui, bien que moins rentables, n’en sont pas moins nécessaires. Je me permets d’attirer votre attention, monsieur le ministre, sur cette proposition. Par ailleurs, diverses missions parlementaires et les travaux de Victor Castanet ont montré, depuis le scandale Orpea, l’opacité des activités des Ehpad privés commerciaux.

à l’effort de prise en charge des personnes âgées dépendantes. Pour toutes ces raisons, le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires soutient pleinement la proposition de loi visant à mettre à contribution les Ehpad privés commerciaux réalisant des profits excessifs. La

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je tiens à mon tour à remercier mon collègue Jean Luc Fichet,

ci prévoit, dans son article unique, la création d’un nouveau prélèvement obligatoire dont les recettes seraient versées à la CNSA, sous la forme d’une contribution additionnelle à la charge de certains Ehpad. Cette dernière serait assise sur le montant d’impôt sur les sociétés acquitté par les gestionnaires les gestionnaires d’Ehpad commerciaux. Son taux serait fixé à 20 % lorsque la rentabilité financière de l’entreprise, mesurée par le rapport entre le résultat net et les capitaux propres, est comprise entre 10 % et 15 % ; il serait fixé à 30 % lorsque ladite rentabilité est supérieure à 15 %.

la simple raison que la population française est inscrite dans une trajectoire de vieillissement tendanciel, laquelle va s’accentuer au cours de la prochaine décennie du fait de l’importance des classes d’âge issues du. Cette évolution démographique se traduira, en matière de politiques publiques de prise en charge de la dépendance, par un accroissement massif des besoins d’investissement dans les Ehpad, estimé à plus de 7 milliards d’euros à l’horizon 2030, et ce alors que la France est plongée dans un contexte qui fait peser des contraintes budgétaires durables sur les finances publiques, locales comme sociales. Je rappelle que cela fait plus de six ans que nous attendons du Président de la République qu’il tienne sa promesse : annoncer enfin le dépôt d’un projet de loi visant à répondre aux défis du vieillissement. est espéré par toutes les parties prenantes, les Français et leur famille comme les professionnels des secteurs de la santé, du social et du médico social. Voilà six ans que les gouvernements successifs nous présentent des écrans de fumée, ce qui engendre légitimement frustration et colère. L’examen, ces derniers mois, de la proposition de loi portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir en France avait permis de souligner la nécessité d’adopter une loi de programmation pluriannuelle pour le grand âge, dotée d’une trajectoire financière,

Comme je l’ai moi même indiqué dans le rapport d’information relatif à l’adaptation du bloc communal au vieillissement de la population, que j’ai présenté la semaine dernière avec mon collègue Laurent Burgoa au nom de la délégation aux collectivités territoriales, il y a pourtant urgence à préparer la société à la massification du vieillissement,

nous à tous ces élus qui n’ont plus les moyens de faire fonctionner leur établissement, donc d’héberger des personnes âgées dépendantes dans les meilleures conditions, et qui font face de surcroît à des problèmes de personnel

rien ne se passe, alors que nous pourrions réinstaurer un équilibre entre Ehpad publics, Ehpad privés à but non lucratif et Ehpad privés à but lucratif en taxant les superprofits de ces derniers. Pour obvier à l’invisibilisation de nos aînés, une planification méthodique et le vote de moyens dédiés s’imposent. Gardons tous à l’esprit que le vieillissement ne signifie pas la fin de la vie. Les personnes âgées ont besoin d’un hébergement et d’un accompagnement adaptés pour vieillir dignement. Si j’osais, je dirais que nous tous ici compterons, un jour,

appellent des moyens d’ampleur. C’est pourquoi, mes chers collègues, je vous invite à voter en faveur de cette proposition de loi, comme le fera évidemment le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain. La parole

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le vieillissement de la population française est un fait de société dont nos politiques publiques n’ont, pendant trop longtemps, pas pris la mesure. Pourtant, le, l’allongement de la durée de vie de notre population et la baisse de la natalité sont connus de tous depuis des décennies. Il n’empêche que s’occuper avec dignité et respect de nos aînés et des personnes souffrant de handicap est notre devoir. nous le savons déjà, nous allons, dans les années à venir, manquer cruellement de places en Ehpad pour satisfaire totalement les besoins de la population, dans la mesure où nous n’aurons pas anticipé cette situation. Je suis moi même président bénévole d’un Ehpad associatif privé à but non lucratif

Quelles sont les dispositions contenues dans cette proposition de loi pour faire face aux retentissantes et scandaleuses affaires qu’a connues le secteur ? Davantage de formation et d’accompagnement des professionnels ? Davantage d’investissement public pour augmenter la capacité d’accueil des Ehpad ? Davantage de contrôles pour déceler à la source les quelques comportements condamnés par toute la profession

taxer davantage n’aura pour effets que de désinciter les Ehpad à investir, d’affecter la qualité des soins dont nos parents ont besoin et, peut être – malheureusement –, de faire augmenter les tarifs de certains Ehpad.

point de vue. Si nous devons revoir notre politique du grand âge et du handicap, faisons le en parlant de formation du personnel, de coût de l’hébergement en Ehpad et d’isolement des résidents, mais ne commençons peut être pas par taxer. Vous l’aurez compris, mes chers collègues,

cette proposition de loi de nos collègues du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain a pour objet la création, pour les Ehpad commerciaux, d’une contribution additionnelle à l’impôt sur les sociétés.

Cette contribution serait de 20 % du montant de l’impôt quand le résultat financier de l’Ehpad est compris entre 10 % et 15 % du montant de ses capitaux propres, ce qui porterait le taux d’imposition sur les bénéfices de 25 % à 30 %. Si le résultat est supérieur à 15 %, le taux de cette contribution additionnelle serait de 30 %, soit un taux d’imposition porté de 25 % à 32,5 %. Notre commission des finances, sur proposition de notre rapporteur Bruno Belin, dont je tiens à saluer la qualité du rapport, s’est opposée à cette nouvelle taxe, estimant qu’elle serait contre productive – cet argument a déjà été largement exposé. Le groupe Les Républicains partage la position de la commission des finances et rejettera donc le texte. Les besoins en places d’hébergement en Ehpad vont exploser ces prochaines années : ils devraient passer d’environ 600 000 actuellement à 700 000 en 2030 et à plus de 900 000 en 2050.

l’utilité de cette taxe assez limitée dans le contexte actuel : aucun Ehpad commercial ne serait vraisemblablement taxé, car aucun n’est suffisamment rentable. Pour toutes ces raisons, je le répète, le groupe Les Républicains, conformément à la position de notre commission, votera contre ce texte. Bien sûr, par delà la question dont il nous est proposé de débattre, la situation des Ehpad, de tous les Ehpad, est plus que préoccupante dans notre pays. Elle nécessite des moyens considérables que seule une réforme en profondeur du financement de la dépendance peut permettre de mobiliser. Des propositions sont sur la table, comme l’instauration d’une deuxième journée de solidarité. La démographie est têtue et la procrastination dans laquelle nous sommes enfermés depuis bientôt quinze ans sur ce sujet est une faute. La discussion est une faute. La discussion générale est close. La commission n’ayant pas élaboré de texte, nous passons à la discussion de l’article unique de la proposition de loi initiale. Sur l’article unique constituant l’ensemble de la proposition

vote. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, il s’agit là d’un sujet éminemment sérieux.

Comme on le constate dans d’autres domaines, ces établissements à but lucratif peuvent présenter des comptes à l’équilibre, voire en déficit, alors qu’ils bénéficient très largement de l’argent public, de l’argent de la sécurité sociale et de l’argent des départements.

parole ?… Je mets aux voix l’article unique constituant l’ensemble de la proposition de loi visant à mettre à contribution les Ehpad privés à but lucratif réalisant des profits excessifs. J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant du groupe Les Républicains. Il va être

Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, la proposition de loi qui est soumise au Sénat aujourd’hui, après avoir été examinée par la commission des lois selon la procédure de législation en commission, traite d’un sujet aride, mais essentiel sur le plan opérationnel, à savoir le mécanisme de purge des nullités. L’actualité le montre : les nullités peuvent avoir des effets dévastateurs sur une procédure, et leurs conséquences sont d’autant plus lourdes qu’elles sont découvertes tardivement. La presse évoquait, encore récemment, le cas de personnes accusées de se livrer au trafic de drogue qui ont été libérées en raison de nullités affectant leur placement en détention provisoire. Certes, il est parfaitement logique dans un État de droit que les vices graves de procédure se traduisent par l’annulation de l’acte concerné, mais il est tout aussi indispensable d’assurer la bonne administration de la justice en évitant les recours dilatoires ou les annulations prononcées au dernier moment. C’est pour concilier ces deux objectifs apparemment contradictoires que le législateur a mis en place, dès le début des années 1990, des outils visant à purger les nullités. Ils s’appliquent notamment dans le cadre des procédures d’information judiciaire puisque celles ci permettent aux parties de soulever les nullités devant le juge d’instruction tout au long de ses investigations. En contrepartie, l’ordonnance de renvoi de l’affaire devant une juridiction de jugement couvre toutes les nullités antérieures à la clôture de l’instruction. Cette pratique peut paraître marginale dans un contexte où les informations judiciaires représentent moins de 2 % du total des dossiers qui passent devant le tribunal correctionnel. Ce sont toutefois les affaires les plus graves, les plus techniques ou ou les plus complexes qui sont concernées – je pense, par exemple, aux « gros » dossiers de narcotrafic, ou encore à la délinquance économique et financière –, si bien que le sujet de la purge des nullités est tout sauf anecdotique. Ces rappels étant faits, j’en arrive à la proposition de loi qui nous occupe aujourd’hui. Déposé par Philippe Bonnecarrère et François Noël Buffet en juin 2024, le texte trouve son origine dans une censure prononcée par le Conseil constitutionnel le 28 septembre 2023 à la suite d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) sur la purge des nullités en matière correctionnelle. En pratique, le requérant avait découvert une cause potentielle de nullité après la clôture de l’instruction, alors même que le vice supposé s’était produit pendant l’instruction elle même : ainsi, la purge était intervenue sans qu’il ait eu l’occasion de faire valoir ses arguments. Le Conseil constitutionnel a estimé qu’une telle situation « méconnaissait le droit à un recours juridictionnel effectif et les droits de la défense » et qu’il appartenait au législateur de prévoir des exceptions à la purge des nullités « dans le cas où le prévenu n’aurait pu avoir connaissance de l’irrégularité éventuelle d’un acte ou d’un élément de la procédure que postérieurement à la clôture de l’instruction ». C’est ainsi que le Conseil constitutionnel a censuré une partie de l’article 385 du code de procédure pénale, en reportant l’effet de cette abrogation au 1 octobre Or, faute pour le législateur d’avoir pu modifier la loi en temps utile, il n’y a plus, depuis cette date, de purge des nullités devant les tribunaux correctionnels. Il nous appartient d’agir sans tarder pour combler cette lacune ; c’est ce que nous permet la présente proposition de loi. Comme son intitulé l’indique, ce texte s’attache à sécuriser le mécanisme de purge des nullités dans l’ensemble de notre droit, et pas seulement en matière correctionnelle : on ne peut que s’en réjouir. Concrètement, la proposition de loi prévoit d’exclure du mécanisme de purge des nullités tous les vices de procédure que les parties ne pouvaient pas connaître avant la clôture de l’instruction, ce qui répond directement à la décision du Conseil constitutionnel. Il est proposé d’appliquer ce principe non seulement à la matière correctionnelle, mais aussi dans les domaines contraventionnel aussi dans les domaines contraventionnel et criminel. Globalement, le texte constitue une réponse pertinente et équilibrée à la censure prononcée par le juge constitutionnel : nous en avons donc préservé l’économie générale. Pour autant, nous avons souhaité apporter des correctifs sur deux sujets, grâce à des amendements que j’ai déposés et qui ont été adoptés par la commission avec l’assentiment du Gouvernement. Ces amendements visent, notamment, à préciser que l’ignorance de la personne mise en cause pour un délit ne peut lui profiter qu’en l’absence de manœuvre ou de négligence c’est une reprise de ce que nous avons prévu, depuis 2021, dans le domaine criminel, et c’est la retranscription d’un principe consacré par la jurisprudence de la Cour de cassation. Ces amendements sont venus, par ailleurs, recentrer la gestion des nullités sur les juridictions du fond. En effet, le texte initial de la proposition de loi créait involontairement des ambiguïtés ou des doublons en confiant cette compétence à la fois au juge du fond et aux chambres de l’instruction ou à leur président, ce qui n’était pas opportun pour la lisibilité de notre droit. Mais, surtout, cela créait également un risque d’engorgement des juridictions d’instruction, déjà bien chargées. C’est pourquoi nous avons simplifié le dispositif et prévu que les juridictions du fond, et elles seules, seraient compétentes pour connaître des nullités que les parties ne pouvaient pas connaître avant la clôture de l’instruction : il me semble qu’il s’agit là d’une mesure de bonne administration de la justice. Pour conclure, mes chers collègues, je me félicite que le Sénat prenne ses responsabilités en adoptant une proposition de loi urgente et nécessaire. Cet état d’esprit s’est exprimé en commission le texte a été adopté dans un climat de large consensus, et je tiens à vous en remercier. Monsieur le garde des sceaux, je vous l’ai dit lors de notre réunion : j’en appelle au Gouvernement pour assurer l’adoption rapide du texte par l’Assemblée nationale. Les juridictions nous regardent, elles attendent avec impatience que nous puissions agir

Monsieur le président, monsieur le président de la commission des finances, monsieur le rapporteur, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs,

Dans sa décision, le Conseil constitutionnel a jugé que le mécanisme de purge des nullités devant le tribunal correctionnel n’était pas conforme au droit à un recours juridictionnel effectif, ainsi qu’aux droits de la défense. Ce mécanisme encadre en effet le droit, pour les parties, de soulever des nullités au cours de l’information judiciaire, puis devant le tribunal correctionnel. En application de ce principe, aucune nullité relative aux actes de procédure réalisés durant l’information judiciaire ne peut être soulevée à l’audience dès lors que le tribunal a été saisi à l’issue de cette même information judiciaire. Il s’agit de la contrepartie logique de la possibilité donnée aux parties de soulever des nullités au cours de l’information judiciaire : devant le tribunal, les parties ne sont plus recevables à les soulever, puisqu’elles ont la faculté de le faire tout au long de la procédure d’instruction. Le Conseil constitutionnel a toutefois censuré l’article 385 du code de procédure pénale, au motif qu’il ne permettait pas à une partie de soulever une nullité devant le tribunal alors même qu’elle n’avait eu connaissance de cette nullité que postérieurement à la clôture de l’information.

Il apparaît indispensable de rétablir ce mécanisme. C’est précisément l’objet de la proposition de loi, et je tiens, à cet effet, à remercier le Sénat pour la qualité et la rapidité du travail mené au regard de l’échéance prévue par le Conseil constitutionnel. Le mécanisme de purge des nullités est essentiel. Il permet de sécuriser les procédures en cours et de limiter les recours dilatoires, afin d’éviter une remise en cause tardive de la procédure, alors même que les parties disposent du droit de saisir la chambre de l’instruction tout au long de la procédure, et que cette chambre peut également relever d’office tout moyen de nullité à l’occasion de l’examen de la régularité de la procédure. Ce dispositif est d’autant plus nécessaire que, lorsqu’un acte procédural est annulé, tous les actes subséquents le sont également, ce qui peut parfois conduire à l’annulation de pans entiers de dossiers de procédures longues et complexes. Ce mécanisme contribue à comme vous l’avez souligné, madame la rapporteure. Il constitue l’une des spécificités de la procédure d’information judiciaire : il est le corollaire d’un cadre procédural qui accorde une place renforcée au principe du contradictoire, et sécurise davantage les procédures d’instruction que les enquêtes préliminaires ou de flagrance, pour lesquelles le contrôle des nullités ne s’exerce qu’au stade de l’audience de jugement. La proposition de loi rétablit le mécanisme de purge des nullités devant le tribunal correctionnel, tout en ajoutant l’exception résultant de la décision du Conseil constitutionnel, c’est à dire en permettant qu’une nullité puisse toujours être soulevée si la partie n’a pas pu en avoir connaissance avant la clôture de l’instruction. Par cohérence, et au delà de ce que prévoit la décision du Conseil constitutionnel, qui ne porte que sur la matière délictuelle, la proposition de loi prévoit cette possibilité devant l’ensemble des juridictions répressives – cour d’assises, cour criminelle départementale, tribunal de police. Par ailleurs, l’un des trois amendements de Mme la rapporteure adoptés par la commission simplifier les règles relatives à l’examen des moyens de nullité qui n’auraient pas pu être invoqués avant l’expiration des délais faute d’avoir été connus, en le confiant à la juridiction correctionnelle ou criminelle compétente sur le fond de l’affaire concernée. Cette modification simplifie le dispositif tout en assurant au justiciable la possibilité de soulever la nullité d’un acte non couverte par les purges, conformément aux exigences du Conseil constitutionnel. Pour toutes ces raisons, le Gouvernement est favorable à l’adoption de la proposition de loi, telle qu’elle est issue des travaux en commission des lois, et tout est fait, madame la rapporteure,

malgré un contexte contentieux et des requérants atypiques, nous voilà face à un texte qui appelle finalement peu de commentaires sur le fond. Nous comprenons très bien la motivation du Conseil constitutionnel qui a conduit à la censure du mécanisme de purge des nullités. Comme l’ont souligné les orateurs précédents, l’article 385 du code de procédure pénale méconnaissait le droit à un recours juridictionnel effectif, ainsi que les droits de la défense. En effet, il ne prévoyait aucune exception à la purge des nullités dans le cas où un prévenu n’aurait pu avoir connaissance de l’irrégularité que postérieurement à la clôture de l’instruction. Dès lors, il a été nécessaire de censurer le dispositif et, par conséquent, de laisser au législateur le soin d’en penser un nouveau. Pour le faire, cette proposition de loi reprend la solution esquissée par le Conseil constitutionnel. Ainsi, les parties pourraient soulever, en matière correctionnelle, le moyen d’une nullité qui « n’aurait pu être connue antérieurement » à deux périodes alternatives : soit dès l’avis de fin d’information et jusqu’à l’ordonnance de règlement du juge d’instruction ; soit devant le tribunal correctionnel, lorsque la partie n’a pu avoir connaissance de la nullité qu’après la clôture de l’information. Surtout, ce texte retient une rédaction large, visant tous les types de juridictions, afin d’écarter le risque d’une censure ultérieure fondée sur des motifs analogues. Tout ce qui a été établi par notre assemblée, et plus spécifiquement par la commission des lois, va donc dans la bonne direction. Je veux saluer l’initiative sénatoriale de François Noël Buffet et Philippe Bonnecarrère, qui ont saisi l’occasion de s’emparer d’une problématique plutôt aride et peu accessible aux citoyens non juristes. Je veux également dire notre intérêt pour les travaux de notre rapporteure, Isabelle Florennes. Aussi, notre groupe n’a pas d’observation particulière à faire sur ce nouveau dispositif. Nous le voterons sans difficulté. Cela étant,

Combien de procédures pourraient être ainsi fragilisées ? Nous entendons souvent les agacements exprimés à l’encontre du gouvernement des juges en général et du Conseil constitutionnel, qui se substituerait au législateur et à l’exécutif. Cette fois, c’est à notre tour de nous montrer critiques sur nos propres défaillances face à l’action des juridictions. Ce n’est d’ailleurs pas la première fois qu’un tel vide est observé en matière de justice. Je pense, par exemple, à la proposition de loi de notre ancien président Jean Claude Requier, qui visait à compléter les dispositions relatives aux modalités d’incarcération ou de libération à la suite d’une décision de cour d’assises. Dans cet autre cas, il fallait combler une carence après l’adoption d’un projet de loi. Ce n’était pas exactement la même situation, mais le même sentiment en ressortait : celui d’une forme d’oubli, en même temps qu’un calendrier législatif mal agencé. Depuis quelques semaines, nous avons un nouveau gouvernement, au sein duquel figurent

Le mercredi 9 octobre dernier, la commission des lois a examiné, selon la procédure de législation en commission, la proposition de loi visant à sécuriser le mécanisme de purge des nullités. Qu’est ce qu’une nullité en droit ? En matière pénale, dès lors qu’un acte est affecté d’un vice grave de procédure, il peut être déclaré nul, c’est à dire qu’il est interdit de faire référence, dans toute la suite des investigations et du jugement, non seulement à cet acte lui même, mais aussi à l’ensemble des actes associés. C’est pourquoi a été créé un mécanisme visant à purger ces nullités, lequel revient à considérer que toute nullité antérieure à la clôture d’une instruction est couverte par l’ordonnance de renvoi devant une juridiction de jugement. En ce sens, l’article 385 du code de procédure pénale prévoyait que le tribunal correctionnel a qualité pour constater les nullités qui lui sont soumises, « sauf lorsqu’il est saisi par le renvoi ordonné par le juge d’instruction ou la chambre de l’instruction Néanmoins, dans sa décision du 28 septembre 2023, déjà évoquée, le Conseil constitutionnel a censuré la dernière partie de phrase, au motif que cette exception méconnaissait le droit à un recours juridictionnel effectif et les droits de la défense.

depuis cette date, le régime transitoire ayant pris fin, le mécanisme de purge des nullités n’est plus opérant, ce qui représente un réel risque de fragilité procédurale et d’instabilité juridique pour un ensemble d’affaires souvent complexes. Il s’agit, en somme, de préserver la bonne administration de la justice. justice. Le présent texte, déposé par nos anciens collègues François Noël Buffet et Philippe Bonnecarrère, s’attache ainsi à sécuriser le mécanisme de purge des nullités dans l’ensemble de notre droit. Pour ce faire, l’article 1 prévoit d’exclure du mécanisme de purge des nullités tous les vices de procédure que les parties ne pouvaient pas connaître avant la clôture de l’instruction, ce qui répond directement à la décision du Conseil constitutionnel. L’article 2 prévoit l’application du texte en outre mer, ce qui est tout de même la moindre des choses. Alors que la commission des lois a adopté trois amendements de Mme la rapporteure visant à prévenir tout risque de nouvelle censure, le Sénat doit désormais prendre ses responsabilités, en adoptant cette proposition de loi pertinente et équilibrée. Vous l’aurez compris, sans suspense, le groupe Union Centriste

un peu plus d’un an, nous avons aujourd’hui à nous prononcer sur un texte permettant de sécuriser le mécanisme de purge des nullités. Pour revenir sur le contexte de cette décision, rappelons que les sages de la rue de Montpensier avaient été saisis à l’époque par un ancien Premier ministre, pour des motifs que je n’ai pas besoin de rappeler ici. Dans sa décision du 28 septembre 2023, le Conseil constitutionnel avait jugé que le mécanisme de purge des nullités en matière constitutionnelle prévue par l’article 385 du code de procédure pénale n’était pas conforme au droit à un recours juridictionnel effectif et aux droits de la défense. La juridiction constitutionnelle avait alors censuré une partie de cet article, nous donnant un an pour voter une loi afin de corriger les effets de cette abrogation. Le gouvernement précédent ayant tardé à se saisir de ce dossier, il est désormais urgent que nous nous emparions de la question des purges de nullité. La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, socle de notre État de droit, dispose, en son article 16, que « toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution ». ». Découle de ce principe fondateur le droit à un recours juridictionnel effectif et le droit à un procès équitable, droits sur lesquels s’est appuyé le Conseil constitutionnel pour rendre sa décision précitée qui nous pousse à légiférer aujourd’hui. Le Conseil contrôle, en effet, les dispositions législatives déjà en application qui portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution. Il œuvre ainsi au respect de l’État de droit. le mécanisme de purge des nullités est loin d’être anecdotique. Notre État de droit a été acquis par le peuple au moyen de luttes politiques et sociales nous permettant aujourd’hui de connaître des droits fondamentaux protégés et des pouvoirs séparés. Il est important de se battre encore et toujours pour le défendre, pour le protéger, et force est de constater que ce combat demeure d’actualité. Nous voterons naturellement ce texte, soucieux de ne pas mettre à mal nos juridictions déjà abîmées par tant d’années de détérioration, mais nous resterons évidemment vigilants sur la protection de notre État de droit,

de ce mécanisme est utile aujourd’hui. Je veux simplement dire deux choses. La première est que le législateur avait un an pour résoudre ce problème. Nous nous félicitons que ce soit fait aujourd’hui, mais peut être le Gouvernement aurait il

intervention est, à première vue, anodin, il en dit long sur l’état de notre système judiciaire. Alors que les auteurs de la proposition de loi avaient prévu de laisser aux juridictions d’instruction le soin d’examiner les moyens de nullité dans certains cas, l’un des amendements l’un des amendements adoptés assigne cette responsabilité à la juridiction compétente au fond. Puisque les juridictions d’instruction sont déjà surchargées, il est impossible de leur assigner cette compétence, explique l’exposé des motifs ! Désormais,

ne doit pas être aux coupes budgétaires, bien au contraire ! J’en profite pour saluer l’engagement du garde des sceaux pour obtenir une hausse des crédits du ministère de la justice ; je veux l’assurer du soutien

résulte de la décision rendue en septembre 2023 par le Conseil constitutionnel en réponse à une question prioritaire de constitutionnalité relative au mécanisme dit de purge des nullités en matière correctionnelle. Sans se prononcer sur le fond, le Conseil a en effet décidé de censurer une partie de l’article 385 du code de procédure pénale, considérant qu’il ne pouvait être conforme à la Constitution dès lors qu’il ne permettait pas à la défense de soulever un vice de procédure qu’elle ne pouvait connaître au moment de l’instruction. de l’instruction. Cette décision s’inscrit dans la volonté de renforcer le droit à un recours juridictionnel effectif et à garantir les droits de la défense. Elle permet une meilleure conformité de notre droit avec l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et l’article 13 de la Convention européenne des droits de l’homme

Or le précédent gouvernement ne s’est jamais saisi de ce sujet. Nous le regrettons – vous n’y êtes pour rien, monsieur le garde des sceaux –, car la définition d’un cadre régissant le mécanisme des nullités est indispensable pour sécuriser les procédures judiciaires et les droits de la défense dans les affaires correctionnelles, mais également criminelles ou contraventionnelles. Étant en quelque sorte acculé, à l’approche de la date butoir, le Gouvernement a finalement décidé de soutenir la proposition de loi de nos anciens collègues François Noël Buffet Philippe Bonnecarrère, texte qui proposait de corriger l’inconstitutionnalité du premier alinéa de l’article 385 du code de procédure pénale et de préciser un cadre plus clair et plus contraignant pour soulever les nullités de procédure. Comme pour de nombreux autres textes, la dissolution décidée par le Président de la République a interrompu le processus législatif. Nous sommes donc confrontés à une situation d’urgence, avec la perspective d’un vide juridique qui n’était de toute évidence pas acceptable. La proposition de loi qui nous est présentée apparaît comme une réponse pertinente et adaptée à la décision du Conseil constitutionnel. Elle permet un équilibre entre le droit à un recours juridictionnel effectif,

collègues, permettez moi de saluer le travail de Mme la rapporteure, qui, par ses amendements, a saisi l’opportunité de ce texte de loi pour harmoniser et simplifier le dispositif, en confiant l’examen des vices de procédure à la seule juridiction compétente au fond. Cela s’inscrit dans une volonté de simplification attendue et dans le respect complet de la jurisprudence du Conseil constitutionnel. La présente proposition de loi doit permettre de limiter les abus procéduraux, d’encadrer plus strictement les délais pour invoquer les nullités et de normaliser les irrégularités sans porter atteinte aux droits fondamentaux des justiciables. Il est en effet indispensable de sécuriser les décisions de justice et le droit des victimes, tout en garantissant des procédures rapides et justes.

dans un esprit de responsabilité et d’efficacité, en souhaitant, monsieur le garde des sceaux, que nous puissions avancer rapidement dans l’aboutissement de cette proposition de loi particulièrement bienvenue.

que la procédure pénale : de 2008 à 2022, le code de procédure pénale est passé de 1 700 articles à 2 400. L’accumulation de petites réformes successives finit, hélas ! par nuire à la cohérence de l’ensemble. Cette inflation s’accompagne également d’une complexité croissante des procédures. Nous devons à nos concitoyens, particulièrement à ceux qui y sont confrontés, de simplifier ce code. La refonte du code de procédure pénale devient de plus en plus urgente à mesure qu’elle se fait attendre. Les États généraux de la justice insistaient déjà sur la nécessité de conduire une étude d’impact sur la faisabilité et l’opportunité de la fusion des cadres d’enquête. Plus largement, nous devons harmoniser et simplifier l’ensemble de la procédure. Tant que ce chantier ne sera pas mené à bien, nous continuerons d’avoir une procédure pénale juridiquement vulnérable et difficilement praticable. Les manquements sont, dès lors, inévitables. La sanction prévue pour les manquements les plus graves à la procédure est la nullité des actes concernés. Ce mécanisme est souvent la cible de vives critiques de nos concitoyens, qui n’acceptent pas que la justice relâche un suspect en raison d’un vice de forme. On peut largement les comprendre ! Les citoyens ont raison de s’indigner : la justice devrait être en mesure de respecter les règles de la procédure. L’État de droit est une nécessité absolue : la justice ne peut pas poursuivre les délinquants qui violent la loi si elle ne s’impose pas à elle même de la respecter. Benjamin Constant disait que « ce qui préserve de l’arbitraire, c’est l’observance des formes ». C’est bien la procédure qui garantit la tenue d’un procès équitable et qui fonde, ainsi, la légitimité de purge des nullités est nécessaire, mais la bonne administration de la justice commande également que les motifs de nullité soient soulevés au plus tôt. Cela permettra à certaines d’entre elles d’être régularisées, si cela est encore possible, ou, à défaut, que les conséquences en soient tirées au plus vite, afin que la justice ne travaille pas en vain. Toutes les parties au procès y ont intérêt. Voilà pourquoi il est prévu que la clôture de la phase de l’instruction purge la procédure des nullités qui n’ont pas été soulevées durant cette phase et qui ne pourront plus l’être ultérieurement. Depuis le 1 octobre – il en ira ainsi jusqu’à la promulgation du présent texte –, notre système pénal ne connaît plus ce mécanisme de purge des nullités en matière correctionnelle. Les justiciables sont donc libres de soulever tous les motifs de nullité, à n’importe quel moment de la procédure, avec tous les inconvénients que cela présente. Les affaires concernées ne sont pas nombreuses, mais elles sont les plus graves ou les plus complexes. La décision du Conseil constitutionnel de septembre 2023, dans la droite ligne de celle de 2021, rappelle que la défense ne peut pas être privée du droit de soulever des motifs de nullité, alors même qu’elle les ignore encore. C’est le caractère équitable du procès qui est en jeu. Il est néanmoins urgent de rétablir le régime de purge, tout en l’adaptant, pour retrouver l’équilibre entre les droits de la défense et la bonne administration de la justice. C’est précisément l’objet de la proposition de loi que nous examinons aujourd’hui. La rédaction retenue par les auteurs, puis améliorée par Mme la rapporteure, est tout à fait satisfaisante. Le texte répond aux exigences constitutionnelles et a le mérite d’uniformiser, autant que faire se peut, le régime de purge des nullités sur ce point. La procédure de législation en commission a démontré son utilité lorsqu’il s’agit d’adopter un texte consensuel et urgent. Le groupe Les Indépendants – République et

Cette proposition de loi intervient à la suite de deux décisions du Conseil constitutionnel portant sur le régime de purge des nullités dans le cadre des procédures correctionnelle et criminelle. Le mécanisme de purge des nullités permet, dans certaines conditions, de rendre irrecevable, devant la juridiction de jugement, toute exception tirée de la nullité de la procédure antérieurement à sa saisine. La purge, qui peut intervenir de manière progressive, durant l’instruction, ou ou globalement, à son terme, permet de stabiliser le dossier à l’approche du procès, en évitant l’invocation tardive et/ou à titre purement dilatoire de nullités procédurales. Plus concrètement, cela signifie que l’ordonnance de mise en accusation « couvre » les éventuels vices de procédure qui lui sont antérieurs. Ce mécanisme, bien que très utile, voire indispensable pour certains dossiers hautement complexes, a été déclaré contraire à la Constitution dans deux décisions récentes du Conseil constitutionnel, fragilisant de nombreuses procédures en cours. En 2021, le Conseil avait une première fois censuré plusieurs dispositions figurant aux articles 181 et 305 1 du code de procédure pénale, au motif que la personne mise en accusation ne pouvait pas contester les irrégularités en cas de défaut d’information sur la procédure criminelle en cours, c’est à dire en cas de défaut de communication d’un acte. Selon le juge, une telle situation portait atteinte aux droits de la défense et au droit au recours juridictionnel. En réaction à cette première censure, le Parlement avait adopté, à la fin de l’année 2021, une procédure légèrement modifiée afin de permettre, dans certains cas limités, l’invocation de la nullité en matière criminelle après le délai normal de purge. la suite d’une décision QPC du Conseil constitutionnel du 28 septembre 2023 relative à la purge des nullités en matière correctionnelle, il est apparu que les garanties offertes par cette exception n’étaient pas suffisantes et ne couvraient pas les cas où la personne intéressée aurait été dans l’incapacité même de connaître, avant la clôture de l’instruction, les informations susceptibles d’avoir une incidence sur la régularité des actes. À l’occasion de cette décision, le juge constitutionnel a censuré les dispositions de l’article 385 du code de procédure pénale permettant la purge des nullités devant le tribunal correctionnel. correctionnel. La proposition de loi vise à tirer les conséquences de ces deux censures, en rétablissant le mécanisme de purge des nullités sous une forme compatible avec la jurisprudence du Conseil constitutionnel. La rédaction retenue est suffisamment large et flexible pour couvrir les différents types de juridictions concernés, afin de régler durablement la question. Il s’agit donc d’un texte opérationnel et efficace, destiné à entrer rapidement en vigueur. Le Conseil constitutionnel avait en effet reporté le plein effet de sa censure d’un an, jusqu’au 1 octobre 2024, date désormais passée. Les circonstances politiques ont malheureusement fait que la présente proposition de loi n’a pu être adoptée de constitutionnalité portées devant le juge constitutionnel pourraient encore faire tomber d’autres pans du régime des nullités. Il est donc essentiel d’agir vite, avant que les effets collatéraux de cette annulation n’endommagent trop de dossiers. Pour conclure, je salue la qualité du travail de perfectionnement du texte initial mené par notre rapporteure, Isabelle Florennes, dans le cadre de la procédure de législation en commission.

Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, la proposition de loi que nous examinons aujourd’hui aborde un sujet technique et fondamental pour le bon fonctionnement de notre justice : le mécanisme de purge des nullités. Bien que le sujet puisse sembler complexe, il revêt une importance cruciale pour la sécurité juridique et le bon déroulement des enquêtes et des procès sur l’ensemble du territoire, y compris dans les outre mer, pris en compte par le texte pour en Il s’agit ici de trouver un équilibre entre la protection des droits de la défense et la nécessité de clore les procédures judiciaires dans des délais raisonnables. Il est aujourd’hui impératif de légiférer de nouveau, car, depuis le 1octobre 2024, il n’existe plus de mécanisme de purge des nullités en matière correctionnelle. Et cela va plus loin

Ce dispositif s’appliquera non seulement en matière correctionnelle, mais aussi aux domaines contraventionnel et criminel, pour couvrir l’ensemble des contentieux concernés. plus détaillée, le texte prévoit que les tribunaux de police, les tribunaux correctionnels et les cours d’assises seront compétents pour examiner ces nullités dans leur domaine respectif, tout en garantissant une procédure simplifiée et conforme aux exigences constitutionnelles. Le mécanisme proposé est donc à la fois équilibré et adapté aux exigences de notre temps. Les ajustements techniques qui ont été apportés en commission de clarifier certaines dispositions, notamment pour ce qui concerne l’application dans les collectivités d’outre mer ou encore pour éviter des chevauchements de compétences entre les juridictions. L’objectif est de simplifier le dispositif tout en assurant son efficacité. Mes chers collègues, ce texte est une réponse nécessaire à la décision du Conseil constitutionnel, et son adoption permettra de restaurer la stabilité de nos procédures judiciaires. Urgent et essentiel, il répond aux répond aux impératifs de justice, dans le respect des droits des parties. Je salue le travail réalisé au Sénat et j’exhorte le Gouvernement et le Parlement à adopter promptement ce texte. texte. Le groupe RDPI se prononcera en faveur de cette proposition de loi, car il est de notre responsabilité d’agir et de s’accorder au profit du bon fonctionnement de nos juridictions. Je mets aux voix,

L’examen de la proposition de loi déposée par notre collègue Jean Michel Arnaud nous offre l’occasion historique de clore ce chapitre et de rendre enfin leur liberté aux communes dans la gestion de l’eau et de l’assainissement, conformément à la position constamment défendue par le Sénat. L’évolution du contexte politique, dont attestent les récentes déclarations du Premier ministre dans cet hémicycle, nous permet d’envisager la reconstruction d’une relation de confiance que l’intercommunalisation forcée des compétences « eau » et « assainissement » avait fragilisée. En tant que conseiller municipal d’une petite commune de 215 habitants et conseiller d’une communauté de communes de 5 200 habitants, dont j’ai également été le président, je mesure combien, dans nos territoires ruraux et de montagne, ce sujet suscite inquiétude et incompréhension. En effet, les attentes des élus locaux sur le terrain nous obligent : l’échéance du 1 janvier 2026, date à compter de laquelle doit intervenir le transfert obligatoire des compétences, approche à grands pas. Plus que jamais, nous avons le devoir d’apporter une réponse sans équivoque à leurs inquiétudes légitimes. C’est dans cette perspective que s’est placée la commission des lois pour conduire ses travaux sur ce texte, travaux qui ont débuté il y a plus de débuté il y a plus de quatre mois. Vous l’aurez compris, je partage pleinement l’objectif exprimé par le texte de Jean Michel Arnaud : il nous faut redonner de la souplesse aux communes, qui sont les mieux placées pour juger de l’échelle la plus pertinente pour l’exercice des compétences « eau » et « assainissement Permettez moi, mes chers collègues, de rappeler quelques éléments de contexte de ce dossier. En matière d’eau et d’assainissement, le Gouvernement a brutalement remis en cause la liberté des communes par le biais de simples amendements déposés à l’Assemblée nationale lors de l’examen du projet de loi NOTRe en 2015. L’objectif était de rendre obligatoire le transfert de ces compétences aux communautés de communes et d’agglomération, à l’instar de ce qui était déjà prévu pour les communautés urbaines et les métropoles. Consciente des difficultés que cette obligation de transfert allait causer aux communes rurales et de montagne, notre assemblée s’y était alors opposée, et elle avait obtenu, en commission mixte paritaire, un report au 1 janvier 2020.

dite loi Engagement et Proximité, a créé un mécanisme très encadré de subdélégation, permettant aux communautés de communes de déléguer les compétences « eau » et « assainissement » à une commune membre ou à un syndicat infracommunautaire, à condition que ce syndicat simplification de l’action publique locale, a apporté un assouplissement supplémentaire en permettant le maintien par principe des syndicats infracommunautaires existant lors de la prise de compétence de l’intercommunalité au 1 janvier 2026. les assouplissements successifs consentis pour atténuer les effets d’un transfert obligatoire imposé aux communes, en méconnaissance des réalités du terrain, ont conduit à une situation d’une grande complexité. Les associations d’élus m’ont notamment fait part de l’incompréhension et de la confusion suscitées par les conventions de délégation. Le risque d’une augmentation de la facture pour les usagers, l’affaiblissement du lien entre le maire et ses administrés, la nécessité de maintenir une fine connaissance des réseaux existants

ne souhaitant pas exercer ces compétences et de communes désireuses de préserver une gestion au plus proche des réalités de leur territoire démontre, s’il le fallait encore, le non sens que constitue ce transfert obligatoire dont l’échéance est désormais très proche. Si le cadre législatif n’évolue pas, le transfert des compétences aura lieu le 1 janvier 2026, avec d’importantes conséquences pour les 3 600 communes qui exercent seules les compétences et les syndicats de communes, qui seront obligés de recourir à une subdélégation défaillante. La proposition de loi que nous examinons repose sur deux principaux axes. L’article 1 vise à créer une dérogation au bénéfice des communes membres d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération située en zone de montagne. Pour ces intercommunalités, les compétences « eau » et « assainissement » redeviendraient facultatives et les communes ayant déjà transféré les compétences pourraient en obtenir la restitution. Pour les communes membres d’une communauté de communes dont le territoire n’est pas situé en zone de montagne, le transfert des compétences « eau » et « assainissement » demeurerait obligatoire, mais serait assorti de nouveaux assouplissements, prévus aux articles 2 et 3. le texte rendrait possible la création de nouveaux syndicats et remplacerait l’obligation de transfert à l’intercommunalité par une obligation de mutualisation des compétences dans des structures syndicales. l’article 4 vise à étendre les possibilités d’intervention des départements en matière de gestion et d’approvisionnement en eau potable, afin de faciliter une gestion à une échelle dépassant les frontières de l’intercommunalité. Comme je vous l’indiquais en préambule, nous avons mené un intense travail collectif afin de trouver la voie la plus satisfaisante pour nos communes, compte tenu de l’imminence de l’échéance de 2026 et des intentions nouvellement exprimées par le Gouvernement. Je tiens particulièrement à remercier mes collègues Mathieu Darnaud, Jean Michel Arnaud, Cécile Cukierman, Jean Yves Roux, Franck Menonville et Paul Toussaint Parigi pour leur précieuse contribution aux discussions qui ont conduit à la solution d’équilibre que je m’apprête à vous présenter. Ainsi, mes chers collègues, je vous proposerai d’adopter un amendement de réécriture globale de l’article 1 qui repose sur deux piliers. D’une part, les communes qui n’ont pas encore transféré les compétences « eau » et « assainissement » à leur communauté de communes ne seront plus obligées de procéder à ce transfert au 1 janvier 2026. Elles retrouveront leur entière liberté. D’autre part, le dispositif ne permettra pas aux communes qui ont déjà transféré les compétences de revenir en arrière. Les transferts déjà effectués ne seront pas remis en cause. Parallèlement, je vous proposerai un autre amendement visant à organiser un dialogue territorial régulier sur l’exercice sur l’exercice des compétences « eau » et « assainissement » au sein de la CDCI. Redonner leur liberté aux communes n’empêche pas de les accompagner, et de rechercher les meilleures solutions de mutualisation au regard des enjeux de qualité et de quantité d’eau. En somme, mes chers collègues, les orientations que vous propose la commission des lois reposent sur trois principes : la liberté, la stabilité et la responsabilité. La liberté, car le cœur de notre engagement a toujours consisté à faire confiance à l’intelligence locale. Les maires sont les mieux placés pour déterminer l’échelle de mutualisation la plus pertinente. La stabilité, car nous souhaitons clore ce chapitre et prévenir l’émergence des nouveaux contentieux qui risqueraient de naître si nous permettions la remise en cause des transferts déjà effectués.

la loi NOTRe, qui a parfois corseté et uniformisé notre pays sans tenir compte de la diversité de ses territoires et de la nature des sujets. L’injonction très vertueuse de la préservation de la ressource en eau a, pour partie, oublié que celle ci ne s’enferme pas dans un périmètre administratif, mais qu’elle coule au fil des bassins versants. Alors que la loi doit protéger la nature comme les hommes, elle a tenté d’uniformiser la première, voulant à tout prix faire d’un jardin à l’anglaise un jardin à la française. Tirons des leçons de cette erreur, et mettons fin aux lois qui contraignent, obligent et interdisent. Préférons les lois qui assouplissent et facilitent, en ayant comme boussole la confiance en nos élus locaux et en leur sens des responsabilités. Excellent que le Premier ministre a affirmé devant vous, ici, sa volonté de travailler en partenariat avec les parlementaires et les élus locaux, en mettant l’écoute et le dialogue au cœur de celui ci. Ce texte est la preuve que nous joignons les actes aux paroles. Cela fait dix ans, mesdames, messieurs les sénateurs, que les compétences « eau » et « assainissement » ne cessent de faire l’objet de débats nourris, de propositions alternatives et d’échanges entre le Parlement et les gouvernements Si la tension grandissante sur la ressource en eau nous appelle collectivement à une exigence accrue de sécurisation des approvisionnements, au bénéfice de nos agriculteurs, de nos entreprises et de nos concitoyens, elle invite également à un effort inédit d’investissement dans nos infrastructures, afin d’assurer une qualité et une plus grande efficience du service public de l’eau. Face aux enjeux qualitatifs autant que quantitatifs de la ressource en eau, il nous faut conjuguer au mieux liberté et responsabilité de choix pour les communes,

de converger pas à pas vers une position d’équilibre. Je salue également l’excellent travail du rapporteur, avec lequel nous avons pu cheminer dans un esprit de dialogue et d’écoute mutuelle.

Attentif aux retours d’expérience, aux difficultés rencontrées et aux propositions formulées, le Gouvernement entend répondre en conciliant pérennisation des transferts d’ores et déjà effectifs et reconnaissance

Concernant les communautés de communes où le transfert a déjà été effectué, elles pourront, grâce aux amendements portés par le rapporteur, déléguer leurs compétences « eau » et la date de leur création. Cela paraît constituer une solution de bon sens. Aussi, le Gouvernement soutient la réécriture de l’article 1 telle qu’elle a été proposée par le rapporteur Alain qui reprend ces principes et rend facultatif l’exercice de la compétence de gestion de l’eau et de l’assainissement pour les communautés de communes qui n’ont pas encore reçu cette compétence. Concrètement, une commune n’ayant pas transféré cette compétence à sa communauté de communes à la date de la promulgation de cette loi disposera de trois possibilités conserver la compétence à l’échelon municipale ; déléguer ou transférer à un syndicat intercommunal ou supracommunal auquel elle aura librement choisi de participer ; transférer la compétence à la communauté de communes.

Cet espace de discussion, qui ne constitue en aucun cas une instance normative à l’égard des communes, permettra de favoriser les échanges autour de ces enjeux.

Je suis intimement persuadée que l’échange de bonnes pratiques est toujours vertueux et que le partage d’expérience dans un cadre de discussion départemental, notamment sur ces enjeux, est bienvenu. Enfin, la proposition de loi nous invite à nous pencher, à l’article 4, sur la question du mandat de maîtrise d’ouvrage confié au département pour des projets de production, de transport ou de stockage d’eau destinée à la consommation. Le Gouvernement est favorable à ce dispositif, qui illustre la pertinence du rôle du département en appui aux communes, dans un objectif de mutualisation et d’efficacité. Il soutiendra donc cette proposition, dans la rédaction amendée par le sénateur Franck Menonville, que je remercie également, afin d’assurer sa mise en cohérence avec le projet de loi d’orientation agricole. Monsieur le président, monsieur le rapporteur, monsieur l’auteur de la proposition de loi, mesdames, messieurs les sénateurs, je crois vous avoir exposé avec franchise et conviction le choix du Gouvernement d’une position responsable, souple, respectueuse des spécificités de nos territoires et à la hauteur des enjeux de ce sujet si essentiel. Elle est le fruit d’échanges constructifs entre un gouvernement à l’écoute des élus et un Sénat exigeant mais sage.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, le sujet que nous abordons ce jour me tient particulièrement à cœur. Maire d’une commune pendant vingt ans, président d’une communauté de communes et sénateur d’un territoire essentiellement rural et montagneux, j’ai été, comme nombre d’entre vous, le témoin des grandes inquiétudes qu’a suscité

et au chemin parlementaire difficile des précédents textes visant à rendre optionnelle la délégation de cette compétence, il nous est aujourd’hui donné l’occasion, grâce à la proposition de loi de notre collègue Jean Michel Arnaud, Michel Arnaud, d’adapter cette mesure aux réalités concrètes de nos territoires, et de faire entendre la voix des maires en leur laissant le pouvoir de choisir. il est temps de réaffirmer, par là même, que la commune reste l’échelon central de la démocratie locale, de montrer aux élus locaux que leur voix porte lorsqu’ils nous alertent sur les problématiques qui les mettent en grande difficulté et lorsqu’ils défendent l’intérêt final de leurs administrés. S’il n’est pas question de remettre en cause le fait intercommunal, nécessaire à la dynamique territoriale, il s’agit d’apporter de la souplesse et de l’agilité à la mise en œuvre d’une compétence extrêmement technique, dont le transfert à marche forcée dans la ruralité et dans les zones de montagne serait préjudiciable. préjudiciable, d’abord, parce que les communautés de communes regroupent des territoires n’ayant pas les mêmes bassins hydrauliques. Or la mutualisation calquée sur des périmètres inappropriés, loin de favoriser les économies d’échelle, induira, hélas ! des dépenses coûteuses, voire faramineuses, nécessaires à la mise en réseau. Ce serait regrettable alors que les territoires de montagne connaissent aujourd’hui une qualité d’eau remarquable pour un coût modéré. préjudiciable, ensuite, parce que les communes se sont déjà organisées en syndicats, quand cela leur semblait pertinent, pour gérer au mieux la compétence « eau » selon des logiques topographiques, et non au gré des frontières intercommunales. qu’il ferait peser sur le consommateur final un risque réel de surfacturation, induit par les moyens techniques, administratifs et financiers que devront mobiliser les intercommunalités pour la mise en œuvre de cette compétence. Ayant été témoin du transfert de la compétence « déchets », je peux attester qu’à ce jour la facture a été multipliée par quatre pour nos administrés. Nous conviendrons tous qu’à l’heure de la rigueur budgétaire, dans une logique de rationalisation des dépenses publiques et d’inflation généralisée,

Faisons donc confiance aux maires qui, face aux sécheresses répétées, ont encore démontré cet été leur formidable réactivité afin de pourvoir aux besoins en eau des habitants de leurs communes. Faisons confiance aux maires qui, sur mon territoire, ont, du nord au sud – mon collègue Jean Jacques Panunzi vous le confirmera –, voté en défaveur de ce transfert obligatoire. Avançons de manière pragmatique et dépassionnée, loin de toute idéologie, et convenons que la spécificité des situations impose ici de repenser l’action publique locale. Le risque d’une augmentation de la facture pour les usagers, l’affaiblissement du lien entre le maire et ses administrés, la nécessité de maintenir une fine connaissance des réseaux existants, ou encore l’absence de correspondance entre les périmètres intercommunaux et les bassins hydrographiques sont autant d’arguments qui plaident en faveur d’une gestion différenciée de ces compétences. Encore une fois, faisons confiance aux maires, car ils connaissent leur territoire et sont en mesure de faire un choix qui répondra à l’intérêt des citoyens.

loi n’est pas le premier texte sur le sujet. M. Barnier rappelait ainsi que, depuis l’adoption de la loi NOTRe en 2015, « cette question […] est une vraie difficulté, peut être une blessure dans la confiance entre l’exécutif et le Sénat ».

Par respect du principe de subsidiarité, notre groupe juge légitime que des élus puissent choisir librement de mettre en commun, ou non, les compétences « eau » et « assainissement », et décider des modalités de cette mise en commun selon les particularités de leur territoire. de loi démontre que bien légiférer est une question de. Corriger les erreurs et améliorer les dysfonctionnements, en faisant trop peu et trop tard, peut avoir des effets néfastes. Au moment où les finances des collectivités sont en danger du fait de coupes rendues nécessaires par des années de gestion pour le moins hasardeuse, sous la présidence Macron, qu’adviendra t il des charges d’investissement destinées aux infrastructures vieillissantes ? Sur ce point, l’exemple de la Guadeloupe est édifiant.

de connaître la vision du gouvernement Barnier sur l’organisation territoriale de notre pays. Nos collectivités sont en attente de nombreuses évolutions : règles comptables nouvelles, transition écologique, démocratie renouvelée, etc. Notre ancien collègue

hivernales dont la réalité brutale annonce de nouveau des étés difficiles. […] Que l’on se place à l’échelle communale ou intercommunale, le problème demeure le même. Aujourd’hui, la politique de l’eau est sous financée dans une fourchette de 800 millions à 3 milliards, voire 4 milliards d’euros par an. On est loin du compte À la veille de discussions budgétaires qui s’annoncent complexes au vu de l’état des finances publiques, et face au perpétuel argument de la dette, lequel phagocyte toutes les politiques que nous devons mener, nous soutenons un cap clair pour lever les incertitudes qui ont pu mener jusqu’à présent à une inaction certaine. loi, si elle est loin de résoudre le problème de l’eau, est un pas de plus vers la différenciation locale, à condition que celle ci soit adossée à une réelle stratégie nationale de l’eau imposée par la raréfaction

aujourd’hui, comme chaque année ou presque, nous examinons dans cet hémicycle une proposition de loi portant sur les compétences « eau » et « assainissement Ce sujet, à la fois technique et politique, soulève des questions centrales sur l’organisation de nos territoires et la gestion de l’eau, une ressource de plus en plus précieuse et stratégique. Permettez moi de commencer par rappeler le contexte. La loi NOTRe du 7 août 2015 a rendu obligatoire le transfert des compétences « eau » et « assainissement » aux communautés de communes et d’agglomération, suscitant

obligatoire pour certaines intercommunalités. Ce report offrait une souplesse nécessaire pour tenir compte des spécificités locales. De même, la loi Engagement et Proximité de 2019 a introduit un mécanisme de délégation partielle de ces compétences aux communes ou syndicats existants. Ces ajustements, qui avaient reçu notre soutien, visaient à renforcer la proximité et l’efficacité de la gestion de ces compétences, sans pour autant revenir sur leur caractère obligatoire. Aujourd’hui, nous sommes invités à examiner une nouvelle proposition d’assouplissement. Nous voyons bien que cette proposition suscite un intérêt certain, tant sur le fond que sur la forme. En témoignent les déclarations récentes, faites ici même, du Premier ministre et l’engagement de la procédure accélérée. Mes chers collègues, nous sommes ouverts aux adaptations, mais nous ne souhaitons pas défaire l’architecture de la loi NOTRe. La gestion intercommunale des compétences « eau » et « assainissement » reste un modèle efficace pour répondre aux enjeux financiers et techniques liés à cette gestion. Nous l’avons dit à plusieurs reprises, et l’avons prouvé au travers de nos différents votes : des adaptations aux réalités locales sont nécessaires, mais il ne peut être question de revenir en arrière. Ce texte appelle aujourd’hui à aller plus loin dans la décentralisation de ces compétences, notamment en zone de montagne où les spécificités géographiques et démographiques nécessitent des ajustements supplémentaires. Notre groupe entend ces préoccupations, mais nous devons veiller à ne pas ouvrir la porte à une remise en cause généralisée des acquis. En effet, nous considérons que les dérogations au transfert de ces compétences ne doivent pas entraîner un détricotage du dispositif. Nous préférons ajuster de manière mesurée, comme cela a été fait jusqu’à présent, à l’article 1. Nous prenons note de l’amendement du rapporteur, lequel ne revient pas sur les transferts de compétences déjà effectués par nombre de communes. Néanmoins, la possibilité laissée à toutes les communes qui n’ont pas encore transféré ces compétences de le faire, en excluant celles qui n’ont pas fait l’usage de la minorité de blocage pour reporter le transfert en 2026, constitue selon nous une atteinte au principe d’égalité devant la loi, principe constitutionnel applicable aux collectivités territoriales et centre de gravité de la souveraineté interne de l’État. Par ailleurs, nous saluons la possibilité accordée aux départements de jouer un rôle plus actif dans les politiques locales de l’eau. Cette disposition, qui découle des travaux de la mission d’information sénatoriale sur la gestion durable de l’eau et reprend en fait le dispositif de l’article 5 de la proposition de loi visant à faciliter une gestion durable et apaisée de l’eau, portée par notre collègue Hervé Gillé, est particulièrement pertinente dans le contexte de raréfaction des ressources et des défis climatiques auxquels nous faisons face. Mes chers collègues, il est temps de prendre de la hauteur. Le transfert des compétences « eau » et « assainissement » ne se limite pas au petit cycle de l’eau ; il faut envisager aussi le grand cycle de l’eau. Il s’inscrit dans une vision globale où nous devons articuler la gestion des ressources en tenant compte des enjeux environnementaux. Face aux défis posés par le réchauffement climatique – les sécheresses, les incendies –, la gestion de cette ressource est devenue une priorité pour nos territoires. Elle implique une responsabilité collective, et il est de notre devoir d’assurer une gestion cohérente, au niveau tant local qu’intercommunal et départemental. Ne sous estimons pas les conséquences d’un mauvais encadrement de cette compétence Je tiens à rappeler que dans l’ensemble des 170 services au taux de rendement le plus faible, 116 sont des services communaux, et donc non mutualisés. La mise en commun des ressources dans certaines zones géographiques est plus que jamais nécessaire ; je pense aux zones montagneuses, qui sont directement confrontées aux enjeux climatiques.

La question de l’ingénierie territoriale est au centre des préoccupations des élus. Vous le savez, les coûts liés à cette compétence ne peuvent pas être supportés individuellement. Les investissements nécessaires pour entretenir et moderniser nos réseaux d’eau sont colossaux. Cela demande une gestion mutualisée. C’est pourquoi nous devons conserver une approche globale intercommunale. Il est important de rappeler que, selon les dernières données, 50 % des intercommunalités exercent déjà la compétence « eau », couvrant plus de 80 % de la population française.

incarnant une réelle dynamique intercommunale qui s’affirme d’année en année. Seulement 14 % des communes appartenant à une communauté de communes exercent encore la compétence « eau » sans aucune forme de mutualisation

que ces ajustements se font dans le respect de l’intérêt général, sans remettre en cause les principes qui ont déjà fait leurs preuves. Nous devons veiller à ne pas déstabiliser un dispositif qui fonctionne bien dans la majorité des territoires. Les élus ont plus que jamais besoin de stabilité au regard des récentes annonces budgétaires… En conclusion, je nous invite à rester fermes sur le maintien du cadre intercommunal, qui garantit la cohérence de notre action en matière de gestion de l’eau. Accompagnons nos intercommunalités dans le développement d’une ingénierie ambitieuse, plutôt que de repousser sans cesse une échéance à laquelle ces établissements publics ont déjà répondu présent. C’est dans cet esprit de responsabilité que notre groupe aborde cette proposition de loi, et c’est pour cette raison que nous ne la soutiendrons pas majoritairement. La parole

Parce que la gestion de l’eau et celle de l’assainissement sont deux compétences fondamentales pour les communes, et que leur organisation doit être optimale. La loi NOTRe affichait certes des objectifs tout à fait louables

La première, c’est que cette loi n’a pas respecté le principe fondamental de libre administration des collectivités territoriales, en contraignant les élus locaux, lesquels étaient largement opposés à cette mesure

Risque d’un affaiblissement de la connaissance des réseaux, absence d’identité entre le périmètre hydrique des communes et celui de l’intercommunalité, possibilité d’une augmentation des tarifs

Nous ne souhaitons pas empêcher les communes et les intercommunalités qui le souhaitent de procéder au transfert de compétences, mais nous ne voulons pas non plus les y contraindre. Nous voulons une solution pragmatique et réaliste, qui laisse le choix, la liberté, à ceux qui connaissent le mieux le terrain : les élus locaux. C’est pourquoi notre groupe s’est profondément réjoui de l’annonce du Premier ministre Michel Barnier de revenir sur le caractère obligatoire du transfert de compétences. C’est la preuve que les élus locaux ont enfin été entendus

Toutefois, elle ne vise que les communes situées en zone de montagne. Une telle exception nous paraît difficilement justifiable vis à vis de toutes les autres communes, que nous, ici au Sénat, représentons. Par conséquent, nous voterons

nous sommes réunis pour discuter d’un sujet les concernant, à savoir la gestion des compétences « eau » et « assainissement ». Lorsqu’on échange avec les élus locaux, les maires, force est de constater que l’eau, cette ressource vitale, est au cœur de nombreuses préoccupations. Il suffit d’observer les conséquences du dérèglement climatique : l’évolution de la pluviométrie conduit à la multiplication et à l’intensification d’épisodes de sécheresse ou d’inondations.

Autant de raisons qui expliquent pourquoi, en matière de gestion de l’eau et d’assainissement, la mutualisation des moyens techniques et financiers peut se révéler stratégique et bénéfique tant pour nos concitoyens que pour les élus locaux. L’article 64 de la loi NOTRe a rendu obligatoire le transfert des compétences « eau » et « assainissement » des communes vers les communautés de communes, en fixant une date limite au 1 janvier 2020.

2026. Pourquoi la loi devrait elle contraindre et forcer les communes à transférer leurs compétences ? Alors que les élus locaux souhaitent davantage de liberté et de différenciation, pourquoi ce transfert devrait il demeurer obligatoire, alors qu’il ne l’était pas avant l’entrée en vigueur de la loi NOTRe ?

Dans le même esprit que le vôtre, monsieur le rapporteur, il me paraît important de permettre à toutes les communes membres d’une communauté de communes qui n’ont pas encore transféré leurs compétences à l’intercommunalité d’en conserver l’exercice. Ainsi, ces communes pourront librement choisir soit de continuer à exercer seules ces compétences, soit de les confier, en tout ou partie, à un syndicat ou à leur communauté de communes. Par ailleurs, je ne suis pas convaincu de la pertinence d’une rétroactivité des transferts

Concrètement, les communes qui n’ont pas fait usage de leur minorité de blocage pour reporter le transfert des compétences au 1 janvier 2026 ne pourront pas obtenir la restitution des compétences. Il en va de même pour les agglomérations.

février, jour de la marmotte dans une petite ville rurale de Pennsylvanie, Phil Connors, interprété par Bill Murray, se retrouve piégé dans une boucle temporelle. Chaque matin, son réveil sonne et il revit toujours la même journée, jusqu’à devenir fou de ne pas savoir comment s’en sortir.

Nous sommes sans cesse alertés par des municipalités, qui s’opposent des motions et des délibérations à ce qui est perçu comme une délégation de compétences beaucoup trop technocratique. Il semble donc absolument nécessaire de revenir une nouvelle fois sur ce dispositif rigide,

s’agit évidemment d’une grande satisfaction, mais nous attendons de connaître les modalités précises d’application de cette annonce. Michel Barnier le sait, les montagnards sont pragmatiques. À ce titre, madame la ministre, sentez vous libre de vous inspirer de nos plus récents

est assurément le cas pour l’eau et l’assainissement, tant les enjeux qui les concernent sont vitaux, qu’il s’agisse de santé publique, d’environnement ou de préservation d’une ressource naturelle toujours plus rare et fragile.

Nous pensons, à l’inverse, que pour déterminer le bon périmètre de gestion des services il faut tenir compte de la diversité des territoires, de leur géographie, des bassins de vie et plus encore des bassins versants. Il faut

Nous connaissons le sens de l’engagement, du service public et des responsabilités des maires. Mes chers collègues, ne les dépossédons pas de ces prérogatives, alors qu’ils sont les mieux placés, sur le terrain, pour déterminer la bonne échelle de gestion et de mutualisation

Dans la vie législative, nous ne le savons que trop, de simples amendements peuvent avoir une immense portée. En 2015, c’est en effet par un simple amendement gouvernemental au funeste projet de loi NOTRe, NOTRe, sans étude d’impact ni avis préalable du Conseil d’État, que le gouvernement d’alors avait fait adopter le transfert obligatoire des compétences « eau » et « assainissement » aux EPCI, y compris dans les communautés de communes.

En effet, ce résultat ne résout pas le problème de fond : la loi oblige toujours les communes à transférer l’eau et l’assainissement à leur communauté de communes au 1 janvier 2026. La mise en place de cette communautarisation généralisée a été voulue, nous dit on, pour éviter une trop forte dispersion des modalités d’exercice de ces compétences, celle ci étant supposée engendrer un manque de rationalisation des services, selon les législateurs de l’époque. La loi NOTRe se donnait ainsi pour objectif une mutualisation efficace des moyens techniques et financiers nécessaires à une meilleure maîtrise des réseaux de distribution d’eau potable et d’assainissement, notamment dans les zones rurales. Nous y voilà, les mots magiques sont lâchés : rationalisation, maîtrise, mutualisation ! Combien d’inepties, mes chers collègues, débouchant invariablement sur de l’incurie en matière de gestion d’argent public, ont été inventées sur la base de ce mirage ? Comment un principe aussi général peut il être opérant, au vu de la très grande hétérogénéité des situations locales ? À l’évidence, la fixation du niveau d’exercice de ces compétences ne saurait être uniforme et déconnectée du terrain ; elle doit, au contraire, relever de considérations matérielles et techniques propres à chaque territoire. Fort heureusement, ici même, le 9 octobre dernier, Michel Barnier, nouveau Premier ministre au parcours d’élu local éprouvé et particulièrement robuste, a déclaré

peut être une blessure dans la confiance entre le Gouvernement et le Sénat. Je salue donc la sagesse de ces propos et la vôtre, madame la ministre, vous qui avez longtemps

succéder à la tribune ! Il ne s’agit donc pas d’opposer les collectivités entre elles, mais de rappeler le principe de subsidiarité, qui doit permettre aux communes de décider du niveau d’exercice de leurs compétences. La parole est à M.

Pernot. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, c’est jour de fête au Sénat ! La demande des maires, relayée par de nombreux sénateurs, va aboutir aujourd’hui l’adhésion à un groupement pour la gestion de l’eau et de l’assainissement va devenir facultative, elle ne sera plus obligatoire ni en 2026 ni plus tard.

ancrée dans la mission du maire ; voilà pourquoi la loi imposant des regroupements était considérée comme un signe de défiance, comme une mesure insultante. L’histoire de la gestion de l’eau a donné naissance à une multitude de situations individuelles très locales dont une mutualisation autoritaire aurait certainement altéré la qualité, la structure accueillante héritant d’une complexité ne pouvant être gérée efficacement à marche forcée. C’est pourquoi il faut rendre grâce à tous les sénateurs qui, déjà conscients de ces difficultés, ont reporté l’exécution des premiers textes de 2020 à 2026. C’est pourquoi il faut également saluer la belle écoute de notre Premier ministre Michel Barnier, qui a promis en ces lieux, lors de la séance des questions au Gouvernement du 9 octobre 2024 – qui deviendra une date anniversaire, n’en doutons pas ! –, que la liberté pour les communes serait maintenant la règle en termes de gestion de l’eau et de l’assainissement. L’adoption de ce texte sera un signal fort à destination de nos collectivités, qui attestera d’une volonté nouvelle d’organiser notre vie publique de manière plus respectueuse, moins verticale et plus partenariale. C’est de cette manière qu’il nous faudra œuvrer pour accompagner les communes, les communautés de communes et les syndicats à relever les nouveaux défis nés de la raréfaction de la ressource. Il convient donc de laisser les territoires s’organiser librement, d’acter, de favoriser, d’inciter, d’inventer des collaborations entre eux, lesquelles devront être les plus circonstanciées possible afin d’obtenir, pour chaque commune, une gestion collective ou autonome idéale des compétences « eau » et « assainissement ». L’ampleur de la mission nécessite des solidarités d’ingénierie, de financement et de moyens en général. L’État, les préfectures et les agences de l’eau, avec les départements, avec les départements, doit se tenir réellement aux côtés des intervenants locaux dans un acte de décentralisation moderne et pertinent pour assurer à chaque citoyen une ressource pérenne, qualitative et quantitative en eau. La réussite de cet objectif passe par une confiance retrouvée entre tous les acteurs. Le vote de cette proposition de loi est une première étape ; elle fait souffler un vent de liberté pour la vie publique locale.

La discussion générale est close. La commission n’ayant pas élaboré de texte, nous passons à la discussion des articles de la proposition de loi initiale. La parole est

Le Sénat a l’occasion de corriger une injustice qui dure depuis plusieurs années et qui se décline en trois volets. Premièrement, une injustice démocratique liée à une erreur de jugement originelle qui a grandement entamé la confiance de nos élus locaux dans toutes les régions de France. Dans mon département de l’Ardèche, comme dans tant d’autres, plusieurs réalités coexistent. Tandis que beaucoup se sont résignés face à la contrainte du transfert, au moins quatre vingt dix communes souhaitent encore rester libres de prendre la décision de conserver ou non les compétences « eau » et « assainissement Une injustice géographique, deuxièmement, liée aux spécificités territoriales de chaque commune. Certaines, bien que limitrophes, ne sont pas situées sur le même bassin versant. D’autres ne peuvent tout simplement pas exercer la compétence

Enfin, quelques unes souhaitent transférer intégralement les deux compétences. Toutes les communes doivent ainsi pouvoir bénéficier d’une plus grande souplesse dans leur gestion, car, au delà de la compétence communale, des préoccupations quotidiennes transparaissent : le coût de l’eau, la disponibilité de la ressource et sa distribution à nos concitoyens. La troisième injustice, enfin, est écologique, face aux sécheresses à venir, plus récurrentes et plus violentes. Soyons réalistes : l’échelon d’exercice des compétences « eau » et « assainissement » ne peut être tranché que localement, en fonction des besoins de chaque commune. Ce texte nous offre ainsi la meilleure opportunité depuis l’adoption de la loi NOTRe de corriger ces trois injustices. Il consacre un pas décisif vers plus de liberté communale. permet enfin le retour à une gestion différenciée et offre à chaque commune la possibilité de trancher définitivement cette question. Pour toutes ces raisons, nous devons soutenir cette proposition de loi sans réserve. La parole

loi en est un bel exemple. Elle traite, évidemment, d’eau et d’assainissement, mais son histoire et ses conséquences débordent nettement le seul périmètre aquatique. Il s’agit ici d’une certaine idée

Nulle obligation, mais nul empêchement. De nombreuses intercommunalités ont déjà franchi le pas du transfert, certaines s’y apprêtent, mais beaucoup

Les grandes régions, les méga cantons, les intercommunalités XXL ou les syndicats géants ont ils conduit à optimiser l’action publique ?

Son objectif était de parvenir à un compromis avec le précédent gouvernement pour assouplir les modalités du transfert des compétences et revenir sur son caractère obligatoire pour les communes de montagne. Le texte aurait dû être examiné après la dissolution de l’Assemblée nationale : il est important de le rappeler pour pour comprendre le contexte de sa rédaction initiale. Il s’agissait pour nous, signataires de cette proposition de loi, d’être pragmatiques et de trouver le chemin pour aller aussi loin que possible dans le cadre qui existait alors. Les annonces du nouveau Premier ministre changent la donne et nous permettent à présent d’espérer aller bien plus loin, jusqu’au retour à un caractère facultatif du transfert des compétences « eau » et « assainissement » pour les communes qui ne l’ont pas encore opéré.

S’il est vrai que la gestion de la ressource en eau constitue un enjeu primordial pour notre avenir et que cela nécessite de la coopération et de la solidarité, c’est, à mon sens, le libre choix des communes qui permettra d’aboutir à des solutions de mutualisation choisie, cohérentes avec la réalité des territoires et des bassins versants. Loin des postures caricaturales, beaucoup d’élus y réfléchissent concrètement. Certains d’entre eux étudient des mutualisations entre bassins versants, mais avec une coordination sur toute l’intercommunalité pour garantir le dialogue et une cohérence dans la stratégie d’ensemble ; d’autres envisagent de transférer une des deux compétences, mais pas l’autre ; certains, enfin, conçoivent des outils de coordination intercommunale qui ne s’opposent pas

La déclaration du Premier ministre Michel Barnier sonne le glas de cette hérésie qui témoignait de la méconnaissance du rural, de ses contraintes et de ses réalités. Comme beaucoup d’entre nous, j’applaudis des deux mains sa prise de position, qui doit désormais se traduire au niveau

Plus de sept années ont été nécessaires pour que la raison l’emporte et le Sénat, une fois de plus, s’est montré clairvoyant. Il s’agit d’un changement de cap salutaire pour les communes, pour la ruralité en général, et pour la Corse en particulier : notre île profondément rurale dispose d’un maillage communal aussi dense qu’éparpillé.

Ce texte et les amendements que nous allons examiner constituent une véritable reconnaissance des libertés locales qui vous sont chères, madame la ministre. d’une loi de liberté et de responsabilité pour les élus et les territoires de France. Je tenais donc à saluer votre action, ainsi que le courage politique du Premier ministre. La parole

la proposition de loi de Jean Yves Roux. Nous saluons le retour à une gestion potentiellement différenciée que cette proposition de loi permet, notamment dans nos territoires ruraux et de montagne, que je connais bien.

celui ci tend à sécuriser la gestion de l’eau en étendant la capacité d’intervention des départements. Ainsi, les départements recevront un mandat de maîtrise d’ouvrage

de catastrophes naturelles en moins de neuf mois et qui ne sait plus comment faire. Au delà de l’émotion, il faut donc construire une politique, et je fais confiance au Gouvernement pour trouver des voies de passage. La parole est à Mme Maryse Carrère, vote. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, je tiens tout d’abord à remercier et à saluer notre rapporteur Alain Marc, qui a réalisé un travail

: ce message de liberté est absolument fondamental. Si, dans les intercommunalités où il y a encore des hésitations, les élus veulent faire le choix du transfert intercommunal, ils le pourront.

a distendu le lien entre les maires et leur population. Et ce n’est pas une bonne chose. Elle a aussi eu, comme l’a souligné notre rapporteur, des conséquences très négatives. Les communes qui sont chefs lieux de canton ont été favorisées au détriment des communes rurales.

Mathieu Darnaud l’a rappelé, et le combat que nous avons mené pendant toutes ces années produit enfin ses résultats, aujourd’hui. Je veux saluer le travail de nos collègues Jean Michel Arnaud, qui s’est battu comme un lion,

Les intempéries de ce jour nous montrent, encore une fois, combien cet enjeu est important. Laissons les maires choisir la solution qui leur semble la plus adaptée et la plus pertinente ! Je ne doute pas du vote de ce soir et vous en remercie par avance,

le rapporteur et, évidemment, par vous même, madame la ministre : nos territoires savent qu’ils peuvent compter sur vous, sur votre engagement et sur votre connaissance fine

Mes chers collègues, par lettre en date de ce jour, le Gouvernement a demandé l’inscription en premier point de l’ordre du jour du mardi 5 novembre prochain : du projet de loi autorisant projet de loi autorisant l’approbation de l’accord sur la création d’un espace aérien commun entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République d’Arménie, d’autre part, et de l’accord sur la création d’un espace aérien commun entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part du projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d’Indonésie relatif à la coopération dans le domaine de la défense ; du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, autorisant accélérée, autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l’État indépendant de Papouasie Nouvelle Guinée relatif à la coopération en matière de défense et au statut des forces du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, autorisant la ratification de l’accord se rapportant à la convention des Nations unies sur le droit de la mer et portant sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale. Ces projets de loi seraient examinés selon la procédure d’examen simplifié. Le Gouvernement a également demandé l’inscription en avant dernier point de l’ordre du jour du mardi 5 novembre, sous réserve de leur dépôt, des conclusions de la commission mixte paritaire sur la proposition de loi visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l’échelle locale. Acte est donné de ces demandes. Nous pourrions en conséquence prévoir de siéger le soir du mardi 5 novembre ; fixer le délai limite de demande de retour à la procédure normale pour l’examen des quatre conventions en forme simplifiée au jeudi 31 octobre à

de la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, visant à poursuivre l’expérimentation relative au travail à temps partagé aux fins d’employabilité. Acte est donné de cette demande. Nous pourrions en conséquence prévoir de siéger éventuellement le soir du mercredi fixer le délai limite de dépôt des amendements de séance sur cette proposition de loi au lundi 4 novembre à douze heures ; et fixer le délai limite d’inscription des orateurs dans la discussion générale sur ce texte au mardi 5 novembre à quinze heures. Y a t il des oppositions ?